J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de commissions mixtes paritaires chargées d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi pour une école de la confiance, sur le projet de loi portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés,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

pour répondre aux besoins de santé de notre population. Retrouvons de la sérénité dans nos débats et je suis sûr que le résultat de nos travaux n'en sera que plus fructueux. ! Acte vous est

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, il ne me semble pas que mon ton habituel dans cet hémicycle nuise à la sérénité des débats.

au mieux dans une dizaine d'années. Or pendant que nous préparons l'avenir, l'urgence est là, autour de nous, dans ces services en grève. Il n'y a certes pas de solution unique, avez-vous dit, madame la ministre, mais il y a des solutions qui sont aujourd'hui réclamées par les personnels urgentistes. Ces solutions consistent à mettre un terme

Monsieur le président, je souhaite faire les rectifications de votes suivantes : concernant les scrutins publics n 130, 132, 133, 134 et 135, Mme Sylviane Noël et M. Daniel Gremillet souhaitaient voter pour

voter pour. Acte est donné de ces mises au point. Elles seront publiées au et figureront dans l'analyse politique des scrutins. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé

Le problème de la démographie médicale constitue aujourd'hui l'un des enjeux majeurs pour de nombreux territoires, et par là même, pour un grand nombre de nos concitoyens. La problématique de l'accès aux soins est ainsi l'une des principales préoccupations ressorties du grand débat. Pour tenter de remédier à cette situation, depuis vingt-cinq ans, des mesures incitatives, le plus souvent de nature financière, sont mises en place par les collectivités territoriales et par l'État, mais en vain. par cet amendement, que, à l'issue de sa formation, tout médecin s'installe pour une durée minimale de quatre ans dans un secteur géographique où l'offre de soins est jugée insuffisante par l'agence régionale de santé. Ce dispositif repose sur le principe selon lequel la collectivité nationale attend un acte de solidarité de la part des jeunes médecins : leur installation, pour une durée provisoire, dans un secteur sous-médicalisé. C'est d'ailleurs cette logique qui prévaut déjà pour un certain nombre de formations et pour les contrats d'engagement de service public.

que de demander à un jeune médecin d'aller exercer, pour une durée déterminée, en zone tendue. Cette mesure ne s'appliquerait qu'aux futurs étudiants en médecine qui se destinent à l'exercice libéral. Les étudiants actuels ne seraient pas concernés, car ils se sont engagés dans les études sans avoir connaissance d'une telle obligation. Enfin, pour des raisons d'équité, ce dispositif s'appliquerait également aux titulaires de diplômes étrangers.

Alors même qu'il existe une cartographie relative à l'installation de nombreux corps de métiers tels que les pharmaciens, les notaires ou les agents de la fonction publique, l'installation des médecins sur l'ensemble du territoire national Résultat : des zones sont désertées par la profession. C'est le seul cas ; nous n'avons pas de problème avec les autres professions de santé, je tiens à le rappeler. Une cartographie médicale semble donc nécessaire pour inverser la vapeur de la désertification de certains territoires, dans le but de réduire considérablement la part des 15 % de personnes vivant en métropole dépourvue de médecin traitant, mais aussi pour protéger les pharmacies rurales menacées du fait de cette désertification. Une fois cette cartographie établie et les zones dites tendues ou sous-dotées identifiées-

qu'il choisit, ce à titre expérimental sur cinq ans, pour donner plus de perspectives au dispositif. Madame la ministre, un territoire qui ne peut plus soigner ses habitants est un territoire qui se meurt ! Or je le sais depuis peu, le village de Tuchan, dans l'Aude, un nouveau médecin généraliste, ce qui met un terme à la desserte médicale. Les zones sous-denses représentent aujourd'hui non seulement une urgence sanitaire et une urgence sociale, mais aussi une urgence en termes d'égalité des territoires. Votre texte ne répond pas à la situation dramatique que nous connaissons dans nos communes. Il n'existe pas de solution unique, certes, mais il faut disposer d'un éventail de solutions ! De fait- cela a déjà été dit -, les mesures incitatives sont malheureusement insuffisantes et la situation empire Parce que le droit à la santé et l'égal accès de tous aux soins doivent nous guider dans ce débat, il est temps d'instaurer sans délai des mesures plus régulatrices, sans doute plus contraignantes, car nous n'avons plus le choix

Dans quel métier n'existe-t-il pas de contraintes ? Cela dit, il ne me semble pas injuste de demander aux médecins de s'engager avec nous pour aboutir à une répartition plus harmonieuse sur l'ensemble du sol national. Permettons au moins l'expérimentation de cette mesure ! Ne restons pas frileux, mes chers collègues ! Il faut évaluer les effets de cette préconisation et savoir si elle peut, réellement ou non, être efficiente pour réduire la désertification médicale. Le nombre d'années proposé- trois ans -me paraît adéquat pour permettre à cette

médicale, il vise à instaurer, à titre expérimental, pour une durée cinq ans à partir du 1 juillet 2020, l'obligation pour tout nouveau médecin libéral d'exercer pendant un an dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins, selon la définition des agences régionales de santé. Les modalités précises de la mise en oeuvre de cette mesure sont définies après concertation du Conseil national de l'ordre des médecins et des organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes médecins libéraux. L'incidence de cette expérimentation est évaluée par le ministère chargé de la santé et le Conseil national de l'ordre des médecins dans le cadre de trois rapports communs. Un rapport d'évaluation est publié avant l'entrée en vigueur de la mesure, un autre sortira au plus tard au 1 janvier 2023 et le dernier rapport sera disponible dans les six mois suivant la fin de la période d'expérimentation.

qui ont supprimé les services publics de proximité. Pour changer cela, je le répète, seule une politique globale de revitalisation permettra de résoudre durablement la problématique de l'attractivité des territoires. l'urgence sanitaire nécessite de dépasser les mesures incitatives et d'étendre aux médecins libéraux un dispositif de régulation à l'installation. Un tel mécanisme existe déjà pour plusieurs autres professionnels de santé comme les pharmaciens, les infirmiers, les sages-femmes ou les chirurgiens-dentistes. Notre amendement a été conçu pour tenir compte des particularités des territoires, mais aussi des contraintes des étudiants tout en donnant de la souplesse au dispositif. Nous proposons donc aux territoires volontaires d'expérimenter l'installation pendant deux ans dans les zones sous-dotées. L'article 40 de la Constitution nous empêchant de proposer des mesures financières, une compensation financière, sous forme d'annuités de retraite,

et nombre d'entre eux ont construit une famille. Il me paraît difficile de les obliger à servir dans un autre territoire que celui dans lequel ils ont peut-être déjà bâti leur foyer.

répondre seuls à des problèmes relevant de l'aménagement du territoire dans des zones où ni des écoles ni des services publics élémentaires n'ont été maintenus par l'État- je rejoins sur ce point le groupe CRCE. Selon moi, c'est bien en amont, lors du parcours de formation des étudiants, que nous devons encourager ceux-ci à l'exercice en ambulatoire, notamment en leur faisant découvrir l'exercice en zone sous-dense. Tel est le sens de l'amendement n° 1 rectifié , que nous avons adopté avant-hier soir

Faut-il comprendre que l'exercice en zone sous-dotée constituerait une sanction pour les étudiants les plus mal classés ? Faut-il comprendre que ces zones devraient se contenter des praticiens du plus faible niveau ? Je ne suis pas certain que cela soit le bon message à envoyer ni aux habitants de ces territoires ni aux étudiants en médecine ! Pour l'ensemble de ces raisons,

Nous rappelons à l'ensemble des parlementaires qu'il est nécessaire aux futurs médecins d'avoir une formation de qualité pour bien prendre en charge leurs patients dans l'exercice de leur futur métier. » « Il est inacceptable de brader la formation des futurs médecins pour répondre aux problématiques d'accès aux soins engendrées par des erreurs politiques d'il y a trente

pourquoi pas ? Qu'on le dise tout de suite ! Nous aurons des médecins salariés, des médecins fonctionnaires qui, comme le rappelait M. le rapporteur, devront s'installer dans des zones sous-denses selon des critères qui seront à déterminer. En ce qui me concerne- et je pense que nous sommes nombreux à partager ce point de vue -, je ne souhaite pas la disparition de la médecine libérale. En revanche, si c'est ce que désirent les jeunes médecins, madame la ministre, entamons

Je m'étonne que certains parlementaires s'offusquent de communiqués de presse qui commentent nos décisions. Je ne vois pas pourquoi l'on ne pourrait pas commenter les choix des sénatrices et des sénateurs que nous sommes.

examinons depuis hier des amendements similaires, mais rien n'est fait pour essayer de régler le problème. On n'a plus de médecins traitants, on n'a plus de médecins de ville ! Il ne se passe pas une journée

très en amont à ces sujets s'en sortent progressivement. Je donnais hier l'exemple de l'Aveyron : regardez ce qu'a fait ce département, c'est extraordinaire Dans nos départements, on subit une pénurie de médecins dans les campagnes, mais aussi dans les villes. L'exemple de Laval, qu'évoquait Catherine Deroche, est instructif. Effectivement, nous y avons mis en place une sorte de cabinet éphémère ; il est tenu par des médecins

mais aussi d'un manque d'effectifs. C'est pourquoi, compte tenu de cette sous-démographie médicale, nous sommes réunis aujourd'hui, dans la sérénité

je comprends tout à fait que la discussion dure assez longtemps, car la situation est très inquiétante pour tous les acteurs locaux, notamment, pour tous les responsables et les décideurs qui, sur place, essaient de trouver le moyen de faire venir des médecins. Je pense que l'attractivité du métier de médecin généraliste

la possibilité d'exercer le métier de médecin et qui la retire quand il le faut. Nous aurons beau prendre toutes les mesures contraignantes que nous souhaiterons, jamais nous ne pourrons empêcher un médecin de s'installer à tel ou tel endroit, qu'il soit conventionné ou non.

Les questions complexes ont ceci en commun qu'elles induisent une tentation autoritaire dans la réponse. Je le dis de façon très dépassionnée.

d'accès aux soins des populations. Elle prendrait par ailleurs en compte l'insuffisante professionnalisation dans la formation que l'Ordre des médecins a encore tout récemment relevée dans son analyse de la non-installation des jeunes professionnels

qui connaît la disparition de ses services publics, un très fort taux de chômage et où le mal-être s'exprime par des votes records en direction des partis extrêmes.

qu'il soit possible de résoudre ce problème en obligeant les jeunes générations de médecins à aller travailler là où elles ne le souhaitent pas.

Le scrutin est ouvert.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

Le scrutin est ouvert.

Madame la ministre, mes chers collègues, je suis particulièrement heureux de saluer la présence dans notre tribune d'honneur de Mme Radmila Shekerinska-Jankovska, vice-présidente du Gouvernement et ministre de la défense de la République de Macédoine du Nord. Elle est reçue aujourd'hui par le groupe interparlementaire d'amitié France-Balkans occidentaux du Sénat, représenté notamment par sa présidente, Mme Marta de Cidrac, et son président délégué pour la Macédoine du Nord, M. Arnaud Bazin. Nous formons le voeu d'un renforcement des échanges entre nos deux pays, dont Mme la ministre- grande amie de la France et parfaite francophone -est l'un des acteurs majeurs. Nous lui souhaitons la plus cordiale bienvenue au Sénat et un fructueux séjour à Paris.

: La parole est à M. Cédric Perrin. Cet amendement vise à permettre à un jeune médecin d'exercer pendant une période de deux ans auprès d'un ou plusieurs praticiens installés, ou auprès d'une structure de soins- établissement de proximité, maison de santé, Ehpad, urgences, dans une zone sous-dense, sans être inscrit au tableau de l'Ordre des médecins. Cette phase de post-internat, au cours de laquelle lui seraient accordées des facilités, l'incitera à exercer dans les zones sous-denses, avant de décider, peut-être, de s'y installer véritablement. L'amendement n° 758, présenté

Pour ce faire, il leur serait permis, pendant une période de six mois renouvelable une fois, soit une année au maximum, de travailler à ce titre sans être inscrits au tableau d'un département. Cette disposition pourrait notamment permettre aux jeunes diplômés d'apporter leur renfort à des médecins relevant de départements différents.

La commission des affaires sociales partage évidemment la préoccupation des auteurs de ces deux amendements. Nous devons en effet développer des leviers permettant d'encourager les jeunes praticiens à découvrir l'exercice ambulatoire, notamment dans les zones sous-denses. Il me semble cependant que les statuts de médecin remplaçant, de médecin adjoint ou de médecin assistant qui existent déjà permettent de répondre à cette problématique. Il ne me paraît donc pas opportun de complexifier encore le paysage des différents modes d'exercice ouverts aux médecins en dehors de l'installation régulière, au risque

sur l'article. L'article 5 revoit à juste titre les modalités de recours à l'adjuvat, afin de soulager les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante. Précisons que l'adjuvat présente trois intérêts non négligeables c'est une pratique valorisée et valorisante par son niveau de rémunération, qui s'exerce en supplément, et non à la place du médecin installé, et qui constitue bien sûr une opportunité pour les étudiants de poursuivre une formation professionnalisante sur le terrain. Nos futurs médecins seront ainsi amenés à découvrir un mode d'exercice et des territoires où ils seront susceptibles de s'installer par la suite. Nous en avons discuté hier soir, les dispositifs incitatifs mis en place depuis plusieurs années commencent à porter leurs fruits,

on oublie parfois les autres zones déshéritées que sont les quartiers relevant de la politique de la ville, dont les problèmes d'attractivité des professionnels de santé sont parfois insolubles. L'article procède à une clarification bienvenue du régime juridique de l'adjuvat en le différenciant de celui du remplacement.

L'article 5 vise à permettre l'adjuvat dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins. Le présent amendement tend à permettre également l'exercice dans ces

rectifié. L'article 4 prévoit que l'exercice en tant qu'adjoint d'un médecin puisse être autorisé dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins déterminées par arrêté, en cas d'afflux saisonnier ou exceptionnel de population, mais également dans « l'intérêt de la population, lorsqu'une carence ponctuelle est constatée dans l'offre de soins par le conseil départemental amendement vise à supprimer le mot « ponctuelle », afin d'étendre les possibilités de recours à un médecin adjoint lorsqu'une carence est constatée par le conseil départemental de l'ordre. Aujourd'hui, de nombreuses zones rencontrent des difficultés dans l'accès aux soins et ne sont pas pour autant identifiées comme telles

Les maires, premiers relais des préoccupations de leurs administrés, sont pleinement légitimes pour alerter sur les difficultés d'accès aux soins rencontrées dans leurs territoires et pour proposer des solutions susceptibles de renforcer la présence médicale, notamment

le caractère ponctuel de la carence dans l'offre de soins ouvrant la possibilité de recruter un médecin adjoint, ce qui revient à étendre la troisième condition prévue dans l'article 5 à l'ensemble des situations de carence dans l'offre de soins. Les conditions figurant à l'article 5 pour le recours aux médecins adjoints sont déjà très larges. Il sera possible dans les zones sous-denses, en cas d'afflux exceptionnel de population, ainsi qu'en cas de carence ponctuelle dans l'offre de soins. que nous ne dénaturions ce dispositif en l'ouvrant trop largement à l'ensemble des situations de carence. Si nous voulons que les différents mécanismes permettant de préserver l'offre de soins restent incitatifs, ils doivent demeurer ciblés. Or la rédaction proposée ouvrirait la possibilité de recourir à un médecin adjoint sur l'ensemble du territoire, et pas seulement dans les zones sous-denses : nous priverions ainsi ces zones d'un outil précieux. Je suis donc défavorable à l'ensemble de ces amendements. L'amendement n° 62 rectifié tend, lui, à rapprocher très largement les régimes de l'adjuvat et du remplacement. Pour la même raison- conserver le caractère ciblé des alternatives à l'installation -, je n'y suis pas favorable.

par le Conseil national de l'ordre des médecins prévu par l'article 5. Je n'y suis pas favorable. J'estime qu'il doit subsister un contrôle du Conseil national de l'ordre des médecins pour prévenir les abus et s'assurer de la compétence des candidats au remplacement et à l'adjuvat. tend à ce que les zones sous-denses susceptibles de bénéficier de l'adjuvat soient déterminées non par l'ARS, mais par le biais d'une concertation avec les collectivités territoriales concernées. Il ne me paraît pas opportun d'alourdir la procédure permettant le déclenchement du recours au médecin adjoint, au risque de rendre le dispositif moins incitatif. Il serait en outre curieux, d'un point de vue juridique, de modifier la procédure de détermination des zones sous-denses prévue par l'article L. 1434-4 du code de la santé l'amendement n° 597 vise à affiner la rédaction retenue par la commission des affaires sociales et à préciser que la compétence du maire de la commune pour l'identification des zones marquées par une carence ponctuelle de l'offre de soins est subsidiaire et vaut à titre de proposition, tandis que l'Ordre des médecins conserve une compétence obligatoire. Cela me semble constituer un apport positif

mettre un terme aux difficultés d'accès aux soins dans de nombreux territoires. Afin de répondre pleinement à cet enjeu majeur, l'ensemble des acteurs du système de santé, quel que soit leur statut, doivent pouvoir se mobiliser et bénéficier pour cela des mêmes dispositifs

Quel est l'avis de la commission ? Les établissements de santé ont la possibilité de recruter des médecins par voie contractuelle. Nous ne le savons d'ailleurs que trop puisque c'est ce qui permet le développement de l'intérim hospitalier. Ils ont par ailleurs des internes. Je vous rappelle que le statut de médecin adjoint est ouvert aux étudiants en troisième cycle. Il n'est donc pas nécessaire de leur offrir cette possibilité supplémentaire. La commission demande donc le retrait

Le présent amendement vise à adapter les modalités d'autorisation d'exercice de la médecine pour l'île de Mayotte dans la mesure où la situation sanitaire y est caractérisée par l'absence d'une médecine de ville apte à répondre aux besoins des populations. Cette sous-dotation a entraîné l'embolie du centre hospitalier de Mayotte, qui, à son tour, ne peut plus assurer au mieux l'ensemble de ses missions de service public, à commencer par ses missions de prévention. Afin de juguler cet effet domino, qui aboutit à un engorgement de l'offre de santé à Mayotte, il est nécessaire de traiter le problème dans le bon ordre. Il faut commencer par améliorer l'offre de médecine de ville en autorisant un médecin

Je suis en règle générale opposé à la remise en cause du ciblage des différents dispositifs d'exercice alternatifs à l'installation, dans la mesure où cela risque de dégrader leur caractère incitatif. Il me semble cependant que la question se pose en des termes différents pour le territoire mahorais, où, comme la commission des affaires sociales a eu l'occasion de le constater lors de son déplacement dans l'océan Indien, l'offre de ville est quasiment inexistante. Je m'interroge cependant sur la potentielle portée du dispositif proposé, dans la mesure où il me semble, mon cher collègue, que l'article visé concerne uniquement les étudiants en médecine, et non les jeunes professionnels. Pour l'ensemble de ces raisons, la commission demande l'avis du Gouvernement, auquel elle se rangera. Quel est l'avis du Gouvernement ? Monsieur le sénateur

de mieux accompagner le développement de l'offre de soins sur l'île. Par ailleurs, de nombreuses mesures ont déjà été prises dans le plan d'action pour l'avenir de Mayotte, en particulier le projet de santé mahorais 2018-2022,

éphémère de Pontarlier, un lieu que j'ai visité. Ils doivent s'acquitter une deuxième fois de la CFE. Celle-ci est relativement élevée, puisqu'elle est calculée sur la valeur locative des locaux, alors même qu'ils n'y exercent pas à temps complet et y génèrent donc peu de bénéfices. On peut par ailleurs noter que les possibilités d'exonération existantes, aux mains des collectivités locales, sont à la fois mal ciblées et mal identifiées par ces dernières. Une exonération de CFE, automatique et compensée aux collectivités par l'État, pourrait être accordée aux médecins exerçant à temps partiel dans une zone sous-dense. Le présent amendement a donc pour objet de conférer un caractère automatique à l'exonération de cotisation foncière des entreprises actuellement mentionnée à l'article 1464 D du code général des impôts, dont peuvent bénéficier les médecins et les auxiliaires médicaux s'installant dans une commune de moins de 2 000 habitants, une commune située dans une zone de revitalisation rurale ou une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins, depuis les dispositions introduites à l'article 173 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. Quel

part, nous sommes passés d'un régime d'autorisation à un régime purement déclaratif à l'Ordre des médecins. D'autre part, nous avons prévu des honoraires bonifiés de 25 % pour les professionnels qui ouvrent

Cet amendement a pour objet de permettre aux infirmiers et infirmières de rédiger un certificat de décès. Dans certaines zones aux caractéristiques géographiques et démographiques contraignantes, rurales, montagneuses, ultra-marines ou insulaires, les familles en deuil doivent parfois attendre des heures, voire des jours,

Il est très difficile, notamment dans certaines zones, pour un médecin de se déplacer dans un délai raisonnable, ce qui n'est acceptable ni d'un point de vue administratif ni sur le plan humain. En laissant aux seuls médecins la possibilité de délivrer un certificat de décès, la loi ne tient pas suffisamment compte de l'évolution de notre société et du développement des déserts médicaux. L'article 5 du présent projet de loi permet également aux médecins retraités ainsi qu'aux étudiants en cours de troisième cycle des études de médecine en France d'établir un certificat de décès. Cet amendement vise à instaurer un dispositif plus souple pour tenir compte de ce phénomène qui touche désormais les espaces ruraux, mais aussi certaines villes.

-, de santé publique et de veille sanitaire, l'examen devant permettre de détecter d'éventuelles maladies infectieusesdont la propagation doit être prévenue.

C'est la raison pour laquelle, à l'Assemblée nationale, j'ai soutenu des amendements permettant à des médecins retraités et des internes, sous certaines conditions, de procéder à la délivrance de ce certificat. En commission, nous avons également soutenu la délivrance de ces certificats par les Padhue. Ces mesures devraient permettre de soulager les territoires qui sont en réelle difficulté aujourd'hui et de répondre aux attentes des familles. Cela étant, je ne peux donner un avis favorable à ces amendements. Le certificat de décès est en effet un document médical qui permet,

une mise en bière immédiate dans un cercueil hermétique lorsque le médecin atteste qu'il s'agit d'une fièvre hémorragique virale, ou dans un cercueil fin simple, mais avec interdiction de soins de conservation du corps lors d'une maladie de Creutzfeldt-Jakob, d'une tuberculose active ou d'un état septique grave.

qui doit être reportée sur le certificat. Celle-ci est d'une importance capitale pour la qualité de la veille sanitaire. Je vous rappelle que tous les certificats de décès font l'objet d'un rapport au registre national des décès tenu par l'Inserm, l'Institut national de la santé et Les médecins sont formés pendant leur cursus initial à l'élaboration de ce type de certificats. Pour toutes ces raisons, mais également parce qu'il s'agit d'une obligation déontologique, je souhaite que l'établissement de ces certificats reste un acte médical et qu'il ne soit pas délégué à d'autres professionnels. Enfin, la rémunération de 100 euros

les tensions devaient persister, nous verrons s'il convient de prendre des mesures nouvelles pour répondre aux inquiétudes. Le Gouvernement est par conséquent défavorable à l'ensemble des amendements.

La participation des médecins retraités à l'établissement de certificats de décès est déjà effective, voire organisée dans certains départements, sous l'égide des conseils départementaux de l'ordre des médecins. Dans les discussions autour de l'objet de cet amendement, il a été question de la constitution de listes de médecins volontaires, ou encore de conditions financières favorables. Cependant, le décret annoncé dans le texte ne renvoie pas à ces questions, mais uniquement aux modalités d'établissement du certificat par un médecin retraité. C'est pourquoi je propose de supprimer l'alinéa 3 de l'article Monsieur le rapporteur,

pour la rémunération perçue à ce titre, du régime applicable au cumul emploi-retraite des médecins en zones sous-denses. Cette rémunération ne donnera donc pas lieu au versement de cotisations sociales ». Pouvez-vous, madame la ministre, nous confirmer que telle est bien l'orientation retenue par le Gouvernement ? Quel est du Gouvernement ? Les médecins retraités, même s'ils sont inscrits au tableau du conseil départemental de l'ordre des médecins, ne peuvent pas effectuer la plénitude des actes qu'ils exerçaient lorsqu'ils étaient en activité. Il est donc nécessaire qu'un décret précise les conditions dans lesquelles ils pourront être amenés à établir les certificats de Ce décret précisera notamment les conditions d'exercice et de formation des médecins retraités pour la réalisation de cet acte, ainsi quele lien avec le médecin traitant habituel, afin de déterminer si le décès est inattendu au regard de l'état de santé de la personne. Il est par ailleurs prévu que la rémunération ne donnera pas

? Selon la commission, il n'y a pas de différence objectivable de compétences entre un médecin en exercice, un étudiant en fin de troisième cycle formé aux certificats de décès, un Padhue en fin de parcours de consolidation des compétences et un médecin retraité.

la commission ? Il a semblé à la commission que les précisions demandées par Mme Rossignol, dont plusieurs termes appellent une définition précise, relèvent plutôt du pouvoir réglementaire.

En réalité, en cas de mort inattendue d'un enfant de moins de deux ans, que le décès soit constaté par un médecin de ville ou un médecin hospitalier,

Par ailleurs, des travaux sont en cours dans le cadre de la préparation du pacte pour l'enfance, afin de mettre en oeuvre des mesures pour renforcer l'effectivité de l'application de ces recommandations.

Dans mon département, il est assez courant qu'aucun décès ne puisse être constaté entre minuit et six heures du matin. Madame la ministre, vous aviez réservé un accueil plutôt favorable

Laurence Cohen, sur l'article. Nous aurons l'occasion de développer notre propos lors de l'examen de notre amendement tendant à la suppression de cet article, mais je veux insister sur les deux raisons principales

publique. Comment interpréter l'alinéa 3, qui entend « simplifier et adapter les conditions et les motifs de recrutement » ? Certes, madame la ministre, l'article 6 a pour ambition, comme l'indique le titre du chapitre III susvisé, de renforcer l'attractivité des carrières hospitalières, ce qui est pleinement au coeur des problèmes que vivent les personnels et les établissements de santé. Nous savons que vous êtes actuellement en pleine concertation avec les professionnels concernés pour limiter le recours à l'intérim dans les hôpitaux publics, position que nous soutenons. C'est une nécessité absolue, quand on sait que, déjà en 2013, le coût de l'intérim médical atteignait 500 millions d'euros et que, vraisemblablement, il est quasiment deux Cette dérive est dramatique et c'est un véritable cercle vicieux. Du fait de leurs difficultés à recruter- près de 30 % des postes de praticiens hospitaliers sont actuellement vacants -, les directeurs et directrices d'établissement n'ont pas d'autre choix que de recourir à l'intérim avec des salaires exorbitants, ce qui grève au final les budgets des hôpitaux et entraîne une compétitivité entre les établissements. C'est ce que nous avons entendu dans tous les territoires lors de notre tour de France des hôpitaux et des Ehpad. Madame la ministre, la commission des affaires sociales a pris le soin d'ajouter, dans l'article 6, un objectif qui était jusqu'ici absent : assurer « un meilleur encadrement des écarts de rémunération entre les personnels titulaires et ceux recrutés par contrat ». Pouvez-vous nous dire si la question des salaires sera abordée dans la concertation que vous menez actuellement ? Un récent article du journal laissait entendre que ce n'était pas le cas ... Or, sans aborder cette question, nous ne résoudrons pas celle de la concurrence avec le privé. Il est également impératif de s'attaquer aux conditions de travail des personnels, ne serait-ce qu'en leur accordant des effectifs en nombre. La parole

il entend, d'une part, créer un statut unique de praticien hospitalier pour favoriser l'exercice mixte entre la ville et l'hôpital, d'autre part, simplifier le recrutement de contractuels. Bien sûr, les conditions d'exercice à l'hôpital sont devenues illisibles du fait d'un foisonnement de statuts, dont les distinctions sont inutilement complexes. Ce constat était déjà dressé par la Cour des comptes dans et nous ne nous opposons pas à une simplification. De même, la diversification des activités est une demande des professionnels et nous reconnaissons volontiers qu'elle rendra les carrières plus attractives. Mais nous regrettons que le projet d'ordonnance qui nous est soumis ne décrive que brièvement de grands principes et ne mentionne aucunement des règles d'encadrement pourtant indispensables. En effet, comment s'assurer que votre réforme ne se fera pas au détriment de l'hôpital, si elle se traduit en un désinvestissement des praticiens hospitaliers de leur travail au sein de l'hôpital public au profit de leur activité privée ? Une autorité locale sera-t-elle chargée de la cohérence de l'ensemble, afin de garantir la continuité et la qualité des soins ? Ce sont bien ces impératifs qui sont en jeu et des dispositifs de contrôle doivent être garantis. De la même manière, nous craignons que les mesures de simplification du recrutement des contractuels ne concurrencent le statut de praticien hospitalier. Nous nous réjouissons de l'apport adopté en commission, sur l'initiative du rapporteur, concernant l'encadrement des écarts de salaires entre les titulaires et les contractuels, facteur important d'attractivité et de fidélisation des praticiens à l'hôpital. Vous nous répondrez sans doute que la concertation doit se poursuivre avec les acteurs pour préciser les contours de ces dispositions. Nous ne pouvons que nous y plier, madame la ministre, mais nous souhaiterions avoir des précisions sur les points évoqués avant de nous prononcer. Je suis saisi

L'article 6 habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures en vue de la création d'un statut unique de praticien hospitalier, qui ira de pair avec la suppression du concours. De façon complémentaire, l'article réforme les conditions de recours à l'emploi médical contractuel dans le cadre d'un nouveau contrat. cet article vise à apporter une solution aux difficultés rencontrées par les hôpitaux sur la question du recrutement, il demeure regrettable, sur la forme, qu'une mesure de cette importance soit renvoyée à une ordonnance. En effet, les conditions de l'emploi médical hospitalier constituent un enjeu central pour le devenir des établissements publics de santé. Un tel sujet aurait donc mérité un débat à l'échelon du Parlement. Sur le fond, des professionnels du secteur ont fait part de leurs inquiétudes sur le possible risque d'une nomination des praticiens hospitaliers par les directions d'établissement en lieu et place de la procédure nationale pilotée par le Centre national de gestion. Ils craignent ainsi le développement de recrutements locaux à la discrétion des managers hospitaliers, créant une hiérarchie entre directeurs et praticiens. Par conséquent, la nomination de ces professionnels devrait rester nationale. En effet, bien qu'imparfait, le processus de recrutement actuel est ouvert à tous reconnaît la compétence médicale et la volonté de l'engagement dans le service public qui sont sanctionnées par un examen devant un collège médical de la spécialité. C'est pourquoi, pour des raisons de transparence du processus, le présent amendement vise à supprimer l'article 6 de ce projet de loi. La parole

entre la ville et l'hôpital. L'article 6 prévoit de fluidifier les carrières entre la ville et l'hôpital pour accroître l'attractivité de l'exercice à l'hôpital nous y voyons un signal positif, mais en regardant de plus près, nous nous apercevons que, pour y parvenir, vous prétendez favoriser l'exercice à l'hôpital des professionnels libéraux, Alors que nous parlons depuis plusieurs jours du manque de professionnels libéraux dans les zones sous-denses, vous allez leur demander demain d'exercer, en plus, dans les hôpitaux publics. Il y a une incohérence Encourager l'exercice partagé entre la ville et l'hôpital, pourquoi pas ? Mais il ne faut pas que cela se fasse au détriment de l'activité hospitalière. Cela risque en fait de contribuer à l'hémorragie qui est déjà à l'oeuvre dans le secteur public. Au motif de simplification, vous remplacez les cinq statuts actuels par un statut unique de praticien contractuel. Au passage, vous supprimez le concours, alors même qu'il est le garant de l'égalité de traitement et de l'absence de favoritisme ; nous ne comprenons pas les raisons de ce choix. Vous voulez réformer le statut de la fonction publique ; c'est normal, les choses doivent évoluer avec le temps, mais à condition de veiller à améliorer les conditions de travail, de revaloriser les rémunérations de titulariser les contractuels qui sont déjà trop nombreux. Devant le flou qui entoure cette réforme, nous demandons la suppression de cet article. commission ? La commission préférerait bien entendu que la réforme du statut des praticiens hospitaliers se fasse par voie législative plutôt que par ordonnance et je regrette que le cadre d'habilitation prévu à l'article 6 soit particulièrement vague- j'en ai fait largement état dans mon rapport.

Or nous sommes convenus, en commission et en dépit de nos fortes réserves sur le nombre de renvois aux ordonnances, de nous montrer aussi constructifs que possible dans l'élaboration de la loi.

Je crois que nous sommes tous d'accord sur l'objectif, car chacun est témoin de la difficulté d'attirer les professionnels dans les hôpitaux publics, notamment dans certaines spécialités.

l'article 6 a pour objet de renforcer l'attractivité des carrières médicales hospitalières, en favorisant la diversification des activités de ces professionnels,

: La parole est à Mme Corinne Imbert. Cet amendement vise à étendre les assouplissements prévus par l'article 6 pour faciliter l'emploi de médecins dans les établissements de santé publics aux établissements du secteur privé à but non lucratif. Ainsi, les professionnels médicaux exerçant en établissement privé à but non lucratif auront la possibilité d'exercer leur art de façon comparable aux praticiens hospitaliers.

à M. Bernard Jomier. Madame la ministre, nous souscrivons à votre objectif de lutte contre les dérives de l'intérim et de renforcement de l'attractivité de la carrière hospitalière, mais parallèlement nous sommes également très attachés à développer un cadre statutaire qui garantisse l'exercice de la mission de service public des praticiens hospitaliers. C'est pourquoi nous proposons que l'exercice mixte, que le Gouvernement souhaite consacrer au travers de la création d'un statut unique de praticien hospitalier, se fasse dans le respect de l'interdiction de cumuler une activité à temps plein et une autre activité, afin de ne pas voir apparaître d'autres dérives.

conditions de travail sont nécessaires pour améliorer l'attractivité des carrières hospitalières. D'ailleurs, la commission des affaires sociales a souhaité que l'ordonnance traite de la question de l'encadrement des écarts de rémunération entre les personnels titulaires et contractuels. Par cet amendement, il s'agit de s'assurer de la compatibilité entre activités principale et

de la commission ? La première précision que comporte l'amendement présenté par M. Jomier ne me paraît pas utile, dans la mesure où le Gouvernement a déjà largement annoncé son intention de travailler dans cette direction-

applicable aux fonctionnaires de l'État. Je me demande si cette précision est bien opérante. Cet article comporte en effet de très nombreuses exceptions au principe de non-cumul qui rendent son contournement relativement aisé.

Il pose donc l'interdiction du cumul d'activités ; c'est l'objet de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 que vous souhaitez voir appliquer aux praticiens hospitaliers. Or l'article L. du code de la santé publique prévoit déjà que cet article de la loi précitée est applicable aux personnels médicaux des établissements publics de santé. De ce point de vue, cet amendement est satisfait. La création d'un statut unique de praticien hospitalier n'est pas de nature à remettre en cause ce principe d'interdiction de cumul d'activités de tous les praticiens exerçant dans des établissements publics de santé pour ce qui concerne ceux dont l'exercice est à temps plein. Ces professionnels conserveront par ailleurs la possibilité d'exercer une activité libérale, dont les conditions devront être adaptées pour tenir compte de la création du statut unique de praticien hospitalier et de l'évolution du contexte territorial, notamment pour permettre que cette activité puisse se déployer sur le territoire, éventuellement hors les murs de l'établissement. Il ne sera donc pas possible, pour ces praticiens exerçant à temps plein, de développer une activité mixte hôpital et ville au-delà de leurs obligations de service dans le cadre que je viens de rappeler. Les praticiens qui feront le choix d'exercer à temps partiel pourront, pour leur part, développer un exercice mixte hôpital et ville. C'est précisément ce que nous souhaitons faire pour apporter de nouvelles réponses aux besoins de l'offre de soins et aux attentes de ces praticiens. Je suis sensible à la préoccupation exprimée dans l'exposé des motifs de cet amendement, à savoir que le développement de l'exercice mixte ne doit pas aboutir à des situations individuelles de temps de travail excessif qui seraient de nature à compromettre la sécurité des soins. Les dispositions qui seront arrêtées devront effectivement prendre en compte ce risque, mais je vous confirme que cet amendement est déjà satisfait. C'est pourquoi j'en demande le retrait.

Je vous y sais sensible, madame la ministre, puisque je vous ai déjà interrogée à ce propos lors d'une séance de questions au Gouvernement. il plombe le budget des hôpitaux par des rémunérations excessives, et, d'autre part, il déstabilise le fonctionnement des services, dont la responsabilité incombe de fait, en priorité, aux praticiens non contractuels. Un décret visant à limiter le salaire journalier des intérimaires a été publié. Pour l'instant, il n'y a pas lieu de se réjouir, puisque, de votre aveu même, madame la ministre, il n'a pas encore porté ses fruits. Il est en effet largement contourné par les directeurs d'établissement hospitalier. Se pose aussi la question des écarts de salaire entre praticiens du secteur public et du secteur privé, que nous ne pouvons pas ignorer. Il apparaît primordial de préserver l'hôpital public et son attractivité pour les médecins. L'objet de cet amendement est donc de préciser que la future ordonnance relative aux statuts des personnels hospitaliers s'attachera, notamment, à valoriser les carrières hospitalières et à encadrer les écarts de rémunération.

Je tiens à préciser, toutefois, madame la ministre, que ce nivellement ne doit pas, dans mon esprit, s'effectuer par le bas. Si l'on veut redonner à l'hôpital public ses lettres de noblesse, il faudra très certainement y mettre le prix. L'amendement n° 300, présenté par Mmes Cohen,

prévoit de « simplifier et adapter les conditions et les motifs de recrutement par contrat pour mieux répondre aux besoins des établissements [ ...] et pour faciliter l'intervention des professionnels libéraux à l'hôpital. Cette rédaction nous fait craindre une fragilisation du statut de la fonction publique hospitalière en multipliant les recrutements sous des conditions dérogatoires. L'article 6 s'inscrit dans la continuité de la réforme de la fonction publique que nous examinerons dans quelques jours : plus de contractuels et moins de fonctionnaires. Nous militons, au contraire, pour la titularisation des contractuels, déjà trop nombreux dans la fonction publique hospitalière, car l'hôpital fonctionne aujourd'hui en se reposant sur des personnels au statut dérogatoire- internes, externes, contractuels et intérimaires. Même si votre argumentaire se veut rassurant concernant vos intentions, qui seraient en réalité non pas de généraliser le recours aux contractuels, mais seulement de le rendre moins complexe, nous sommes particulièrement sceptiques. Certes, les formes de contrat pour praticiens hospitaliers sont multiples, avec les statuts de praticien contractuel, de praticien attaché et de praticien attaché associé, de clinicien hospitalier ou de praticien adjoint contractuel. Nous pensons que l'attractivité des établissements est liée non pas au type de contrat, mais à la possibilité de titularisation, aux matériels à disposition, aux effectifs et aux conditions de travail.

comme l'amendement présenté par Mme Imbert, est irrecevable au titre de l'article 38 de la Constitution. Je le répète pour ceux qui n'étaient pas là au moment où je l'ai dit à Mme Imbert, le Parlement ne peut pas

Arnell, le 1° de l'habilitation mentionne déjà, parmi les objectifs visés, le renforcement de l'attractivité des carrières hospitalières et l'encadrement des écarts de rémunération.

l'avenir de l'hôpital public. Dans tous les contacts que nous avons pu avoir avec eux, les directeurs d'établissement ont mis en avant cette faible attractivité de la profession de praticien hospitalier et leurs difficultés à recruter.

de mettre en place des combinaisons entre leurs établissements pour se prêter, en quelque sorte, des praticiens spécialisés, afin de permettre à ceux-ci de bénéficier de statuts particuliers à durée limitée et d'augmenter leurs salaires. Nous touchons également

Cet amendement vise à inscrire dans la loi le principe d'un plan national de santé au travail et de qualité de vie au travail des professionnels hospitaliers. La santé des soignants est un enjeu majeur. Or la qualité de vie au travail des professionnels de santé s'est considérablement dégradée ces dernières années. Ce plan devra traduire l'ambition partagée par le ministère des solidarités et de la santé, la sécurité sociale, les établissements listés à l'article 2 de la loi de 1986, les partenaires sociaux et les grands organismes de prévention de constituer un socle commun pour la promotion de la santé et de la qualité de vie au travail. Cette démarche devra faire l'objet d'un accompagnement méthodologique et financier fort

vise à promouvoir la santé et la qualité de vie au travail, dont nos personnels ont plus que jamais besoin aujourd'hui pour prendre en charge nos patients, dans le contexte difficile que nous connaissons.

ont malheureusement mis en oeuvre des politiques de réduction des dépenses de santé. Ces réductions, que nous avons dénoncées à l'époque, ont eu des conséquences désastreuses sur les conditions de travail des professionnels hospitaliers. Les chiffres le montrent, le mal-être au travail a entraîné de nombreux suicides de personnels. Des rythmes de travail élevés, un manque de moyens matériels,

Ainsi, selon le rapport de recherche sur la santé des soignants, publié en 2018 par le professeur Didier Truchot de l'université de Bourgogne-Franche-Comté, 23 % des soignants ont des difficultés à dormir tous les jours ou presque. Les professions les plus touchées sont les infirmières, 28,8

Les infirmières et les aides-soignantes représentent, de loin, les groupes professionnels les plus frappés par les problèmes de santé. Les professionnels hospitaliers ne peuvent plus travailler dans de telles conditions. Cela n'est plus possible ! Écoutez la chanson des infirmières de Valence ; écoutez les appels de détresse. de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé, nous proposons de reprendre une proposition émanant de la Fédération hospitalière de France, la FHF, visant à élaborer un plan national de santé et qualité de vie au travail des professionnels de santé. Tel est le sens de cet amendement. au travail pour les professionnels de santé du secteur hospitalier. Les conditions de travail et l'assurance d'un suivi médical des professionnels hospitaliers conditionnent en partie l'attractivité de ces métiers. Pour ne donner qu'un exemple, les métiers d'infirmier et d'aide-soignant connaissent aujourd'hui une crise des vocations inédite. Les hôpitaux peinent à pourvoir leurs postes, et les formations sur les territoires ont du mal à se remplir. Si la dégradation des conditions de travail n'en est pas la seule raison, elle y contribue fortement. Par ailleurs, la qualité de vie des praticiens la qualité de vie des praticiens a des conséquences évidentes sur la qualité des soins pour les patients. Il s'agit ici de proposer de recréer un cercle vertueux, des conditions de travail sereines pour les professionnels entraînant des conditions de prise en charge optimales pour les patients. Promouvoir les démarches de qualité au travail nécessite une analyse de l'organisation du travail, afin de s'inscrire dans une logique de prévention et non plus de réparation. Sur le modèle du plan national quadriennal de santé au travail élaboré par le ministère du travail en concertation avec les acteurs de la prévention, le présent amendement vise à inscrire dans la loi le principe d'un plan national. Ce plan est, pour beaucoup de professionnels, une étape indispensable pour renforcer la dynamique de notre système de santé. C'est également un signal fort que nous pouvons envoyer dès aujourd'hui aux professionnels de soins pour leur assurer que leurs conditions de travail sont notre priorité.

dans l'article L. 1411-1 du code de la santé publique, lequel définit la politique de santé de la Nation dans sa globalité, et pas dans ses détails.

A du présent projet de loi prévoit que le projet social de chaque établissement doit intégrer un volet spécifiquement consacré à la qualité de vie au travail des personnels hospitaliers. J'attends

des personnels hospitalo-universitaires qui vont les encadrer. Nous avons déjà discuté de ce problème au début de l'examen de ce projet de loi. Les fortes inégalités territoriales dans l'accès aux études de médecine se retrouvent dans le taux d'encadrement des étudiants en médecine par les enseignants. Le rapport de la Cour des comptes de 2017 sur le rôle des CHU dans l'enseignement supérieur et la recherche médicale a mis en lumière les grandes disparités qui existent dans la répartition des personnels hospitalo-universitaires entre les CHU. Ainsi, en 2015-2016, un poste d'enseignant titulaire ou non titulaire correspondait à 5,29 étudiants à l'université de Paris 5, contre 15 à l'université de Lille 2. Madame la ministre, vous avez répondu à nos collègues députés que la répartition des postes hospitalo-universitaires dépendait du nombre d'étudiants à former. C'est tout à fait exact. J'ajoute qu'il faut aussi prendre en considération la capacité des établissements de santé à faire de la recherche les disciplines pratiquées dans le CHU. Actuellement, de nombreuses universités en région ne disposent pas de postes hospitalo-universitaires titulaires dans toutes les spécialités. Au total, notre système est morcelé et caractérisé par de fortes inégalités de moyens, ce qui compromet l'homogénéité des formations. Notre amendement vise donc à essayer de corriger ces disparités en favorisant une répartition plus équilibrée des personnels titulaires. Quel

tant sur les budgets des hôpitaux que sur l'organisation des services. Son objet est de permettre la non-imposition des heures supplémentaires au-delà du seuil de 5 000 euros annuels en place aujourd'hui. Cette mesure a pour but, à court terme, de favoriser les heures supplémentaires pour les praticiens en poste, et de limiter ainsi, je l'espère, le recours aux contractuels. Si l'on ne peut agir sur le recrutement des praticiens de manière directe, on peut agir sur l'attractivité des métiers, notamment grâce à cette mesure de déplafonnement de l'exonération sur le temps de travail additionnel. Tel est le sens de cet amendement. L'amendement n° 709 rectifié, Bernard Jomier. Il s'agit d'un amendement similaire. Comme nous l'avons déjà indiqué, la commission avait souhaité aborder la question de la rémunération dans le secteur hospitalier à l'article 6, en prévoyant que l'ordonnance traite bien de la question de l'encadrement des écarts de rémunération entre les personnels titulaires et contractuels. et contractuels. Puisque nous partageons cet objectif en matière d'attractivité des carrières hospitalières, en particulier des praticiens hospitaliers, nous vous proposons une mesure en ce sens, de mise en oeuvre et d'efficacité immédiates. Reprenant une proposition de la FHF, notre amendement a pour objet de déplafonner l'exonération en matière de temps de travail additionnel,

d'un chiffrage du coût qu'elle représenterait pour les finances publiques. Je me demande par ailleurs quelle serait l'incidence de cette mesure sur l'intérim, madame Guillotin. Certains intérimaires sont embauchés lors de périodes de congés, et je pense que l'incitation au temps de travail additionnel ne changerait pas grand-chose à de telles configurations. Nous demandons donc une évaluation de la portée de cette mesure au Gouvernement et une analyse de sa pertinence au regard des évolutions engagées dans le cadre de l'article 6. Quel est du Gouvernement ? Si nous partageons évidemment le souhait de rendre plus attractives les carrières et de réduire la part de l'intérim, je rappelle que j'ai déjà pris des mesures visant à mieux encadrer le recours à l'intérim médical, notamment avec un arrêté en En l'occurrence, vous proposez une non-imposition du temps de travail additionnel au-delà d'un plafond de 5 000 euros. Ce plafond correspond à environ seize périodes de temps de travail additionnel. C'est donc une mesure assez positive, car une partie non négligeable du temps de travail additionnel effectué par les praticiens

En effet, il nous paraît impératif d'encadrer et surtout de limiter la concurrence qui existe quand un praticien hospitalier démissionne pour exercer une activité libérale en ville ou bien quand il cumule les deux fonctions.

Ils expliquent qu'ils ne peuvent pas financièrement s'aligner sur les rémunérations existant dans le privé. Si l'on ajoute à cela les conditions de travail difficiles dans les établissements publics, nombre de médecins, toutes spécialités confondues,

des praticiens pour les remplacer. C'est bien la preuve d'un manque d'attractivité, tant du point de vue des rémunérations que des conditions de travail, qui, nous l'avons déjà dénoncé, se dégradent.

Que ce soit pour les praticiennes et praticiens démissionnaires ou pour ceux qui exercent à temps partiel, nous soutenons la proposition faite dans cet article 6 A pour limiter la concurrence directe,

de l'exercice hospitalier et d'amplifier les coopérations entre la ville et l'hôpital. Si ces objectifs ne peuvent qu'être partagés, il convient de se montrer prudent sur les effets de concurrence qui pourraient en résulter au sein d'un territoire, au détriment de l'hôpital public. C'est pourquoi la commission des affaires sociales a proposé de compléter l'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique, qui interdit aux praticiens démissionnaires d'un établissement public d'entrer en concurrence avec cet établissement pendant les deux années qui suivent la fin de leurs fonctions. Elle entend prévoir également une limitation des éventuelles situations de concurrence directe entre les différentes activités des praticiens hospitaliers exerçant à temps non complet.

Cet amendement vise à procéder à plusieurs aménagements rédactionnels de l'article 6 A introduit par la commission des affaires sociales, sans modifier sa portée sur le fond. Il s'agit ainsi de sécuriser le dispositif de prévention des situations de concurrence et de le rendre plus opérationnel.

Dans l'objectif légitime et indispensable d'améliorer l'attractivité des carrières publiques, l'article 6 du présent projet de loi, que nous venons de voter, prévoit d'accorder aux praticiens hospitaliers des hôpitaux publics la possibilité d'exercer également en ville, leur conférant ainsi l'avantage de pouvoir exercer en libéral à la fois en ville et à l'hôpital. En effet, les praticiens hospitaliers du secteur public ont déjà, par ailleurs, le droit d'exercer une activité libérale au sein de leur hôpital, ce qui est interdit aux praticiens du secteur privé non lucratif. Les établissements de santé privés d'intérêt collectif, ou Espic, rencontrent des difficultés pour attirer et fidéliser les médecins dans leurs structures. Dans un certain nombre de cas, leurs praticiens n'ont pas accès aux mêmes opportunités que celles qui existent dans les hôpitaux publics.

doivent donc être accessibles de manière identique à tous les praticiens qui exercent dans les différents types d'établissements composant le service public. Cet amendement vise ainsi à permettre la pratique d'une activité libérale aux praticiens salariés à temps plein des Espic, de la même façon que celle-ci est aujourd'hui autorisée aux praticiens hospitaliers à temps plein des établissements publics de santé. commission ? En l'état actuel du droit, l'activité libérale intra-établissement n'est ouverte qu'aux praticiens statutaires exerçant à plein temps au sein des établissements publics de santé. Ce choix a historiquement été fait en raison du régime encadrant la rémunération des praticiens des hôpitaux publics et des Espic : le statut qui s'applique aux praticiens

d'un statut, les secondes d'une convention collective, laquelle donne beaucoup de souplesse aux contrats. C'est précisément pour tenir compte des contraintes supérieures associées à l'exercice sous statut que la possibilité de réaliser une activité libérale a été historiquement ouverte aux praticiens hospitaliers. De façon plus générale, l'objectif du Gouvernement n'est pas de développer une offre de soins supplémentaires ouvrant le droit à des dépassements d'honoraires ; il est plutôt de favoriser l'accès aux soins. Madame la sénatrice, je vous propose donc de retirer votre amendement ; à défaut, j'y serai défavorable.

Les agences régionales de santé, créées en vertu de la loi HPST, ont pour but d'assurer un pilotage unifié de la santé en région, de mieux répondre aux besoins de la population et d'accroître l'efficacité du système. Le présent amendement vise à les supprimer, compte tenu des résultats plus que moyens

Les ARS supprimées, leurs services et agents seraient replacés sous l'autorité directe du préfet de région, et des préfets de département s'agissant de leurs délégués départementaux, dont ils dépendaient antérieurement. Le lien des élus avec les représentants traditionnels de l'État que sont les préfets s'avère plus adéquat, ceux-ci étant davantage à l'écoute des attentes et des besoins des élus locaux et des territoires. Les parlementaires et les élus locaux sont en effet en contact permanent avec les préfets, alors qu'ils sont

en en confiant la présidence à un élu issu du conseil régional, répondant ainsi à une partie de vos préoccupations. Il ne me semble pas que l'on puisse demander aujourd'hui la suppression des ARS

elles ont su développer une vision globale de la santé intégrant la prévention et la promotion de la santé, ainsi que la santé environnementale ; elles voient la totalité de l'offre de soins, libérale et hospitalière- contrairement aux agences régionales d'hospitalisation qui existaient auparavant -, ainsi que l'offre médico-sociale

pour faire en sorte que les médecins aient envie de s'installer : elles les accompagnent dans leur installation, notamment dans les zones sous-denses, et elles les orientent grâce à des dispositifs incitatifs.

capables de rencontrer les élus dans les délégations territoriales, parce que c'est effectivement en ce domaine que pêche notre capacité à interagir avec vous.

ajoute la « promotion de la santé » aux compétences partagées entre l'État et les collectivités territoriales. En ajoutant la promotion de la santé aux missions des collectivités territoriales, en plus de l'administration, de l'aménagement du territoire, du développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, met, certes, l'accent sur leurs responsabilités en matière de promotion de la santé. Toutefois, au-delà d'une réalité qui peut prendre la forme de contrats avec les ARS sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et l'accompagnement médico-social, cet article ajoute une mission aux collectivités territoriales sans transfert de crédits. Alors que les mesures d'austérité contraignent déjà les collectivités réduire certaines missions de service public, ajouter la promotion de la santé va encore aggraver cette situation, puisqu'elles devront faire davantage avec moins de moyens.

et les collectivités territoriales en matière de « promotion de la santé », ce qui conduit davantage à confirmer ce qui se fait déjà qu'à imposer une charge supplémentaire aux collectivités territoriales. La commission ne voit cependant pas d'obstacle à la suppression de cet article à la portée

impression de discuter d'un projet dont les nombreux éléments ajoutés de manière disparate masquent difficilement un manque de vision cohérente d'ensemble. En second lieu, cette mesure me semble même potentiellement dangereuse, car elle instille de la confusion dans l'organisation de notre système de soins. Alors que le plan Ma santé 2022, au diapason des dernières recommandations du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, conforte la coordination des professionnels de premier et deuxième recours, vous introduisez un nouvel étage

Je crains donc une forme de déstructuration du parcours de santé au détriment,, du patient, et je doute même que les professionnels y comprennent quelque chose et s'en saisissent réellement. Madame la ministre, ce type de dispositions illustre un grand besoin un grand besoin au regard de ce projet de loi, celui de clarifier un schéma prospectif d'ensemble, cohérent, de l'organisation de notre système de soins. Ce dernier

commission ? Je me suis en effet interrogé sur cet article 7 C, qui vient ajouter un nouvel outil à ceux qui existent déjà, à savoir les équipes de soins primaires, les ESP, et les En cela, la création des équipes de soins spécialisés ne participe pas d'une démarche de simplification. Toutefois, tout ce qui peut favoriser la coordination entre les acteurs du système de santé me semble utile. La commission a donc émis un avis défavorable

en prévoyant un triptyque médecin généraliste, pharmacien et infirmier libéral, auquel viennent s'ajouter, selon les besoins des patients, les autres auxiliaires médicaux. L'article L. 1411-11-1 du code de la santé publique prévoit actuellement que l'ESP est composée d'un « ensemble de professionnels de santé ».

n'est pas différenciée de l'approche populationnelle confiée aux CPTS. Les missions des ESP définies dans le code de la santé publique entrent en collision avec celles qui sont confiées aux CPTS : les premières ont pour mission la coordination clinique de proximité, alors que les secondes exercent une mission de coordination au niveau d'un bassin de population sur un territoire. La clarification des missions et de la composition des équipes de soins primaires doit permettre de répondre aux défis du vieillissement de la population et de l'explosion des maladies chroniques. Il est essentiel d'asseoir cette coordination de proximité sur un triptyque qui peut induire un effet systémique sur la prise en charge du patient. Ce triptyque médecin généraliste, pharmacien, infirmier libéral doit être clairement inscrit dans la loi, tout en permettant à d'autres professionnels de santé d'être inclus dans l'ESP, en fonction des spécificités de prise en charge du patient. Quel est l'avis de la commission

Encore une fois, je comprends cette volonté de clarifier et de rappeler quels doivent être les professionnels engagés dans des équipes de soins primaires.

pouvoir s'engager dans ces équipes de soins primaires. Pour autant, à trop normer le dispositif dès le départ, alors que la dynamique de création s'instaure sur le territoire, on risquerait d'être contre-productif. C'est la raison pour laquelle je propose le retrait de cet amendement

Cet amendement vise à demander pourquoi, malgré le décret de 2016, il ne se passe rien, et tend à mettre des moyens à disposition pour expérimenter, pendant trois ans, le développement de cette médecine de proximité et de l'accès aux soins.

de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 compte, parmi ses objectifs, celui de « favoriser la présence de professionnels de santé dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins

Nous souhaitons associer davantage les parlementaires à la politique de santé sur le territoire, en les intégrant aux conseils territoriaux de santé. Les parlementaires sont très fréquemment sollicités sur les questions d'accès à la santé leur participation aux conseils territoriaux de santé leur permettra d'être informés de la situation de l'offre de santé sur le territoire de leur circonscription, d'être davantage associés à la mise en oeuvre effective des projets régionaux de santé dans les territoires Aujourd'hui, les conseils territoriaux de santé contribuent à l'élaboration, à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation des projets régionaux de santé. Ils sont chargés d'identifier les insuffisances en termes d'offre, d'accessibilité, de coordination et de continuité

Sur les conseils territoriaux de santé, je suis beaucoup plus dubitatif. Je trouve que c'est un peu une mesure, disons, d'affichage. Par ailleurs, madame

il faudrait écrire : « les sénateurs ». Je suis un peu méfiante depuis que « quelques députés et quelques sénateurs » siègent dans les instances locales

avec notamment la présence intermittente d'au moins un professionnel de la santé visuelle, orthoptiste ou ophtalmologiste. J'avais déposé des amendements visant à étendre ces contrats à des sites d'exercice secondaire et aux

les conditions d'embauche des orthoptistes par les médecins conventionnés spécialisés en ophtalmologie. Ce décret s'est avéré complexe et désincitatif, puisqu'une seulement de contrats ont été signés, alors que l'étude d'impact de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 tablait sur plusieurs centaines. Par ailleurs,

ont été formés et ont formé les autres médecins de leur établissement à identifier, derrière les symptômes ou les diagnostics apparents que les femmes décrivent lorsqu'elles se présentent, par exemple,

diagnostics. Aujourd'hui, nous sommes sortis des phases expérimentales ou incitatives : il faut prévoir par la loi que tout établissement susceptible d'accueillir des enfants

C'est un enjeu de formation des professionnels plus que de désignation d'un référent unique, lequel n'est pas forcément légitime par rapport à ses collègues. En réalité, nous avons choisi une autre méthode, consistant à responsabiliser les centres de psychotrauma

Entre le projet médical partagé, les projets territoriaux de santé mentale, les contrats locaux de santé et les contrats territoriaux de santé élaborés par les communautés de nous y retrouver ... L'objectif de l'article 7 est donc de simplifier l'existant et de créer des projets territoriaux de santé- PTS -intégrant toutes les actions menées par les différents acteurs d'un même territoire, aussi bien pour la ville que pour le médico-social et l'hôpital. Évidemment, sur le papier, l'idée paraît bonne. Je pense sincèrement que de telles démarches collectives peuvent faire vivre la démocratie sanitaire.

nous sommes un peu sceptiques sur ses effets concrets pour l'amélioration de l'accès aux soins, par exemple. Nous laissons toutefois le bénéfice du doute à ces PTS et faisons confiance à l'intelligence collective des professionnels de santé. C'est dans cet esprit que nous avons déposé

professionnelles territoriales de santé dans l'élaboration des projets territoriaux de santé, en en faisant des acteurs centraux de la démocratie sanitaire. Cette importante bataille pour faire des questions de santé un débat ouvert à tous les citoyens passe également par l'implication des élus. La disposition prévoyant la présence d'un parlementaire a été supprimée- nous venons d'en débattre -, mais les élus sont les représentants des citoyens travaillant dans la proximité. C'est particulièrement le cas des élus municipaux et des conseillers territoriaux qui eux-mêmes travaillent sur ces questions, notamment en ce qui concerne l'âge ou le handicap.

la plus complète possible, il est indispensable que nous disposions d'outils indépendants de mesure et d'évaluation de la santé sur les territoires. Dans le Nord-Pas-de-Calais, l'Observatoire régional de la santé a fermé pour raisons

Nous l'avons dit : cette voie est prometteuse, car elle est une des clés de la structuration d'une offre de première ligne suffisamment robuste pour répondre aux enjeux de la transition démographique et épidémiologique de notre population, et ainsi soulager l'hôpital. Soyons clairs, cet article est largement perfectible : sa rédaction est assez indigeste, et le dispositif ne contribue pas à simplifier un millefeuille que de plus en plus de rapports s'accordent à qualifier de complexe et d'illisible. toutefois l'intérêt de conforter un outil de coordination qui fait progressivement ses preuves, les communautés professionnelles territoriales de santé, fonctionnant selon une approche ascendante qui fait la part belle, pour le moment, à la souplesse et à l'initiative des acteurs de terrain. terrain. Reste que le temps de gestion de projets est aussi du temps médical en moins pour les professionnels. À cet égard, il est dommage que le projet de loi n'évoque pas le rôle que devraient davantage jouer les ARS dans l'accompagnement de ces projets. Sur les missions spécifiques que devraient remplir les CPTS, le choix a été fait de ne pas les préciser dans la loi. Je souhaiterais pourtant rappeler les rôles sur lesquels ces communautés sont attendues, notamment en matière de décloisonnement des secteurs sanitaire et médico-social et de prise en charge ambulatoire.

Dans une seconde phase de maturation, elles devraient être à même d'assurer le maintien à domicile des personnes âgées, l'organisation de la prise en charge de différentes pathologies chroniques liées aux particularités épidémiologiques des différents territoires et de faire de l'éducation thérapeutique à destination de ces patients chroniques-

La fusion des régions a entraîné un éloignement entre les élus locaux et les administrations régionales- c'est un fait. Depuis lors, nous sommes nombreux à rencontrer des difficultés pour faire vivre la relation avec les ARS. Nous avons des difficultés à obtenir des réponses à nos sollicitations, y compris parce que nous ne savons pas toujours à qui nous adresser. Or les difficultés d'accès aux soins préoccupent beaucoup les élus locaux, qui sont en demande de réponses, mais peuvent aussi être force de propositions. Il paraît donc important, sur des sujets aussi sensibles et majeurs que la santé et l'organisation des soins, de renforcer les liens entre élus et ARS. J'insiste donc sur la nécessité d'avoir un référent ou un interlocuteur privilégié dans chaque ARS, lequel serait chargé des relations avec les élus, qui ne se sentent pas toujours écoutés face aux problématiques de santé. La parole

de l'hôpital et du secteur médico-social. Ceux-ci auront la possibilité de constituer des projets territoriaux de santé à leur propre initiative, afin de développer des synergies et des complémentarités entre les soignants de ville, l'hôpital et le médico-social. Ces projets ne seront pas délimités territorialement, mais ils procéderont plutôt de la bonne organisation des parcours de soin. Afin de développer ce mode d'organisation « à la carte », sans pour autant superposer trop d'entités administratives, les acteurs du projet territorial de santé définiront par eux-mêmes le périmètre de leur action. Concernant les communautés professionnelles territoriales de santé, cet article prévoit de les soumettre à l'approbation de l'ARS concernée afin d'assurer la cohérence de ces communautés sur l'ensemble du territoire. Cette mesure nous semble de nature à offrir une meilleure qualité et une meilleure continuité de l'offre de soins. En effet, cela permettra de fluidifier le parcours de soins au travers de la coopération de tous les acteurs de santé des territoires. L'ensemble des professionnels de santé que notre groupe a auditionnés préconisent

Daudigny, sur l'article. L'article 7 porte sur la création des projets territoriaux de santé, avec l'objectif d'éviter le fonctionnement en silos de la médecine de ville, de la médecine hospitalière et des différents établissements médico-sociaux. Répondant aux aspirations des acteurs de santé à mieux coopérer entre eux, l'inscription dans un exercice coordonné constitue un argument décisif pour l'installation des nouvelles générations.

sorte que les acteurs de l'ambulatoire puissent se rencontrer et examiner ensemble les questions de santé populationnelle, apportant ainsi une dimension de service au public issue de l'initiative des acteurs de terrain. Veillons néanmoins à ne pas mettre en place un dispositif au travers duquel le pouvoir administratif des agences régionales de santé s'affirmerait dans toute sa rigidité, sans ménager une place suffisante à l'initiative des professionnels de territoire et à la démocratie sanitaire.

ne doit pas prendre le pas sur cette négociation. Celles-ci ne doivent pas devenir des objets administratifs centrés sur des objectifs trop contraints. Si l'on constate un véritable dynamisme dans la constitution des CPTS- nous avons rencontré, au cours de ces dernières semaines, beaucoup d'acteurs enthousiastes

Il paraît aussi nécessaire de clarifier l'articulation entre les CPTS et d'autres dispositifs de coordination, tels que les plateformes territoriales d'appui, dont le positionnement et la mission ne semblent pas très lisibles.

projet régional de santé et s'assurer de la cohérence de son territoire géographique avec celui des autres CPTS ; ce ne saurait être un examen qui compliquerait la tâche des porteurs de projets. La parole

un PTS commun entre médecine de ville et médecine hospitalière avec les équipes de soins primaires, les CPTS, l'hôpital, le médico-social, les élus. Cet outil aura vocation à veiller à la continuité de l'offre de soins sur l'ensemble du territoire et favorisera les synergies entre les professionnels. Madame le ministre, au travers de ce dispositif, vous avez fait le pari de coordonner l'offre de soins des territoires. Nous saluons cet objectif, qui paraît pertinent

Malgré le fait que l'article 7 est révélateur de l'attente pressante de nos concitoyens quant à l'établissement de projets territoriaux de santé, dans l'objectif de répondre à l'expansion des déserts médicaux, la réponse qu'il apporte ne paraît cependant pas à la hauteur des enjeux. Après les contrats locaux de santé, les conseils territoriaux de santé, les schémas régionaux de santé et autres projets médicaux partagés, rien n'indique que les projets territoriaux de santé trouveront leur place parmi l'éventail déjà disponible de dispositifs administratifs. Pour atteindre une meilleure couverture territoriale en matière de santé, la simplification devrait être d'un meilleur secours que la complexification. Cet amendement vise donc à supprimer cette nouvelle invention administrative.

d'une logique intégratrice. Il faut toutefois, me semble-t-il, laisser les acteurs de terrain s'en saisir, en veillant à conserver la souplesse de l'outil pour rester dans une logique incitative et ne pas en faire une usine à gaz. L'objectif est partagé : c'est celui d'un décloisonnement entre les acteurs de soins de ville, l'hôpital et le médico-social, mesure indispensable pour construire des parcours de santé cohérents pour les patients. Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur la suppression de l'article 7.

L'article 7 institue un projet territorial de santé, qui jouera un rôle de levier en matière de décloisonnement entre les professionnels de santé de ville et les établissements de santé ou acteurs médico-sociaux. Les premiers seront structurés à l'avenir autour de ces PTS, destinés à mailler l'ensemble du territoire. L'article L. 1434-2 du code de la santé publique concerne la constitution du projet régional de santé. Il détermine que le projet régional de santé fixe des objectifs généraux et les résultats attendus à dix ans. Un schéma régional de santé est établi pour cinq ans notamment sur la base d'une évaluation des besoins sanitaires. Il peut être mis en oeuvre par les contrats territoriaux de santé, les contrats territoriaux de santé mentale ou encore les contrats locaux de santé. Toutefois, la loi reste actuellement muette sur la durée de ces trois types de contrats. Par cohérence avec le schéma que ces contrats viennent décliner, cet amendement vise à coordonner leur durée avec celle du schéma régional. Quel est l'avis de

Je ne souhaite pas inscrire dans la loi une durée normative, afin, justement, de laisser cette liberté, cette souplesse, qui favorise la dynamique de terrain et, au contraire, ne la freine pas. C'est pourquoi je suis défavorable à cet amendement.

Notre amendement vise à renforcer la représentation des élus et des usagers au sein des conseils territoriaux de santé, en créant des comités territoriaux des élus. Nous portons ainsi une demande émanant notamment de la Fédération hospitalière de France nous a alertés sur l'insuffisance de la participation des CTS aux prises de décision, sur le manque de capacité d'initiative, d'impulsion et de validation. En outre, elle fait le constat d'une sous-représentation des élus locaux et des usagers au sein des CTS. Aussi, il nous semble indispensable, pour aller dans le sens d'une plus grande démocratie sanitaire, d'associer de manière plus effective les élus et les usagers aux décisions territoriales des politiques de santé. Un renforcement de la participation des élus locaux et des usagers est d'autant plus nécessaire que le projet de loi accentue le mouvement de territorialisation des politiques de santé et de mise en concurrence des établissements de santé. Le droit fondamental à la protection de la santé et l'égal accès de tous nos concitoyens aux soins doivent être garantis. Notre amendement vise à permettre aux représentants des citoyens et aux usagers de s'assurer de la mise en oeuvre effective de ces principes. Quel

les impacts de l'environnement sur la santé doivent être évalués au mieux afin de prévenir divers risques sanitaires dus à la pollution des milieux et aux agents physiques. Les évaluations doivent être réalisées à différentes échelles afin de garantir leur qualité et leur efficacité. C'est pourquoi les conseils territoriaux de santé doivent utiliser au mieux ces évaluations réalisées à l'échelle régionale ou infrarégionale, évaluations dont les données sont au coeur de l'objectif du diagnostic territorial partagé : « Identifier les besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la population sur la base de données d'observation. Ces plans régionaux prennent en compte les facteurs de risques spécifiques aux régions ; ils ont pour objet de mieux prendre en considération les enjeux locaux. Ainsi, ils sont de nature à apporter un savoir essentiel à l'élaboration des diagnostics par les conseils territoriaux de santé. Préciser leur utilisation est nécessaire pour assurer une prise en compte importante de la santé environnementale dans les diagnostics réalisés par les conseils territoriaux de santé, une prise en compte qui ne figure pas aujourd'hui à l'article L. 1434-10 du code de la santé publique. Grâce à une prise en considération des évaluations et des recommandations réalisées par le plan régional de santé environnementale dans l'élaboration des diagnostics, les membres du conseil et les professionnels de santé seront informés et pourront ainsi transmettre les informations aux populations concernées. Cet amendement tend également à s'assurer que les signalements des lanceurs d'alerte sont utilisés. La loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique visait à permettre la protection des lanceurs d'alerte et à définir leur statut. cette avancée, il faut réellement être à l'écoute et tenir compte des signalements, qui ont pour objet de révéler les situations que nous ignorons. La qualité des diagnostics élaborés par les conseils territoriaux ne peut que s'accroître si ces derniers se montrent attentifs aux voix des lanceurs d'alerte.

dans l'Ain, une affaire ancienne ayant refait surface récemment. Les diverses hypothèses mettent en cause des raisons environnementales. Ce cas précis nous démontre l'importance d'avoir une véritable connaissance des risques pour la santé de la situation environnementale des territoires. connaissances sont parfois empiriques, ce qui explique l'importance d'être attentifs aux alertes et connaissances produites par des dispositifs déjà existants. L'objet de cet amendement est d'empêcher que des crises sanitaires se perpétuent ou se développent en agissant à la source des problèmes. De plus, cela encouragerait des actions préventives de la part des professionnels de la santé et des populations.

est beaucoup plus courte, mais plus compréhensible ... Sans nier l'importance des enjeux soulevés, il ne paraît pas nécessaire de mentionner dans la loi toutes les données existantes prises en compte dans le diagnostic territorial partagé. Si nous le faisions, nous

dans l'élaboration des projets territoriaux de santé, en liaison étroite avec les communautés professionnelles territoriales de santé et les établissements et services de santé. Le CTS, qui est une instance de démocratie en santé reconnue et identifiée, permet de rassembler l'ensemble des acteurs de santé dans les territoires. La proposition de Médecins du Monde et de la Fédération des acteurs de la solidarité rejoint notre demande de démocratie sanitaire en partant d'une structure qui existe déjà dans les territoires. S'y exprime le besoin d'une meilleure concertation et d'une meilleure coordination entre les acteurs du parcours de santé.

contribuent à faire avancer la relation avec l'ambulatoire. Il faut mettre en avant les professionnels de santé et non les structures si l'on veut obtenir des projets territoriaux adaptés aux situations locales. L'amendement

L'article 7 prévoit la création du projet territorial de santé et assure l'approbation des CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé, par le directeur général de l'ARS. sanitaires et sociaux, et l'APF France handicap sont à l'origine, vise à garantir une meilleure opérationnalité des projets territoriaux de santé. Nous rappelons que le conseil territorial de santé est l'instance de démocratie en santé qui paraît légitime pour mener à bien cet exercice. Il garantit la représentativité de tous les acteurs d'un territoire et la cohérence avec le diagnostic partagé qu'il a élaboré. La multiplication de collectifs d'acteurs et de projets- équipes de soins primaires, communautés professionnelles territoriales de santé, plateformes territoriales d'appui, conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie, conseils territoriaux de santé -risque d'apporter de la confusion et une déperdition dans la mobilisation des acteurs, en multipliant les instances et groupes de travail, voire de créer de la concurrence entre différents collectifs d'acteurs. Cet amendement prévoit enfin de mettre en place une évaluation périodique des projets territoriaux de santé par le conseil territorial de santé.

Reconnue par l'Organisation mondiale de la santé depuis 1986, la médecine thermale peut jouer un rôle prépondérant dans la prévention de maladies et offre une thérapie complémentaire et alternative aux prescriptions médicamenteuses ainsi qu'aux opérations chirurgicales. Les établissements thermaux entrent dans un cadre de service médical rendu sans avoir d'effets secondaires et sont donc d'un très grand intérêt pour la santé publique. Ils ont, à ce titre, toute leur place dans les projets territoriaux de santé. Leur intégration serait d'autant plus intéressante qu'ils se situent très souvent dans des zones sous-denses et qu'ils ont un effet de structuration dans certains territoires, en particulier les territoires de montagne. Les intégrer à un exercice coordonné serait donc bénéfique tant pour les établissements thermaux que pour les autres professionnels de santé.

que le PTS fixe des objectifs en cohérence avec les besoins de la population. La présente disposition permet de garantir une dynamique autour de ce nouveau dispositif des projets territoriaux de santé en cas d'absence d'initiatives des acteurs. Quel est l'avis de commission ? Concernant les amendements n315 et 515, le conseil territorial de santé sera associé à la démarche et au suivi des projets territoriaux de santé puisqu'il en assurera l'évaluation.

le texte de l'article 7 vise, plus généralement, les établissements et services de santé, sociaux et médico-sociaux, mais rien n'empêchera les établissements d'associer leurs CME à ces démarches d'élaboration des projets territoriaux de santé, dans le cadre de leurs compétences.

les professionnels de santé se saisir d'outils dont la réussite est étroitement conditionnée à leur engagement et à leur volontarisme. Le projet de loi supprime l'initiative de l'ARS en cas de carence d'initiatives des professionnels dans la constitution des CPTS. Gardons la même souplesse s'agissant des PTS. En conséquence, la commission

La méconnaissance des besoins d'accompagnement de ces populations, notamment des migrants, est un facteur de refus de soins. C'est pourquoi il est essentiel que le projet territorial de santé prenne en compte

La permanence des soins est l'une des préoccupations majeures de la population dans les territoires. Si son organisation est prévue par divers dispositifs, il est indispensable que le PTS fixe les modalités d'amélioration de cette permanence qui fait partie intégrante de l'organisation des parcours de santé. Le projet territorial de santé élaboré par les CPTS devra décrire les modalités d'amélioration de l'accès aux soins et de la coordination des parcours de santé. Les patients peuvent rencontrer des difficultés d'accès aux soins, particulièrement lorsqu'il s'agit de soins non programmés. Ces derniers sont parfois à l'origine d'une désorganisation du cabinet médical, mais aussi, et peut-être surtout, d'un engorgement des urgences. Aussi, il importe que le PTS puisse organiser l'accès aux soins non programmés, en tenant compte des spécificités de chaque territoire. Par ailleurs, la politique de dépistage doit également pouvoir être inscrite dans le projet territorial de santé, afin d'en renforcer l'efficacité.

centres et maisons de santé. Or l'organisation de la permanence des soins est jugée aujourd'hui peu visible et peu compréhensible par de nombreuses familles, qui, dès lors, n'ont pas d'autres solutions que de se rendre dans les services d'urgence pour être prises en charge, être prises en charge, ce qui a pour conséquence d'engorger ces services. La référence à la seule amélioration de la continuité des soins ne permet pas d'apporter les réponses adaptées aux familles en matière de soins non programmés. Le projet territorial de santé doit donc définir l'organisation de cette permanence des soins et expliciter clairement les engagements de l'ensemble des acteurs au sein d'un territoire. L'amendement Chasseing. La permanence des soins est l'une des préoccupations majeures de la population. Si son organisation est prévue par divers dispositifs, il est indispensable que le PTS fixe les modalités d'amélioration de cette permanence

n° 209 rectifié. Le projet territorial de santé élaboré par les CPTS devra décrire les modalités d'amélioration de l'accès aux soins et de la coordination des parcours de santé. les patients peuvent rencontrer des difficultés d'accès aux soins, particulièrement lorsqu'il s'agit de soins non programmés. Ces derniers sont parfois à l'origine d'une désorganisation du cabinet médical ou d'un engorgement des urgences. Aussi, il importe que le projet territorial de santé puisse organiser l'accès aux soins non programmés, en tenant compte des spécificités de chaque territoire.

Cet amendement a pour objet d'inscrire dans la loi la participation des établissements publics de santé aux communautés professionnelles territoriales de santé. Cette participation est en effet parfois contestée par les professionnels de ville et les établissements de santé nous ont fait remonter leurs difficultés à intégrer les CPTS.

à prévoir la prise en charge, au sein des PTS, de l'accès aux soins des personnes en situation de handicap, des personnes à mobilité réduite et des personnes en situation de précarité.

dans l'élaboration du diagnostic territorial partagé. Il tend à inscrire la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants dans le contenu de ce projet territorial de santé.

Je regrette d'ailleurs que les conséquences des violences faites aux femmes et aux enfants soient trop souvent sous-estimées. Les troubles psychotraumatiques sont pourtant graves, très graves, fréquents, avec des conséquences durables sur le devenir des victimes. Ils peuvent durer des années, voire une vie entière, si les victimes ne bénéficient pas de soins et d'un suivi important. Et faute de soins ou de suivi,

de la commission ? La commission a recentré le contenu du projet territorial de santé dans le but d'en faire un outil souple à la main des professionnels de terrain, ciblé sur des priorités comme la continuité des soins et la coordination du parcours entre ville, hôpital et médico-social.

En outre, et comme pour les amendements n 524 rectifié et 490 rectifié, il ne paraît pas opportun de mentionner spécifiquement la permanence des soins : celle-ci dispose déjà d'un cadre d'organisation et de planification qui a valeur opposable, à la différence du projet territorial de santé. Il ne faut pas ajouter à la confusion en faisant du PTS un nouvel outil de gestion de la permanence des soins.

les mentionner explicitement permet de mettre l'accent sur des enjeux prioritaires : comme dirait l'autre, cela ne mange pas de pain ! La commission a donc émis un avis favorable

714 rectifié. Sans pour autant nier l'importance des enjeux soulevés, le PTS n'a pas vocation, me semble-t-il, à se substituer à l'ensemble des autres documents et outils existants. Nous n'avons pas besoin d'énumérer dans la loi tous les enjeux que ce projet doit prendre en compte, au risque d'oublier de mentionner certains enjeux importants ou de décourager les initiatives des professionnels de santé.

vais aller un peu dans le même sens. L'articulation ville-hôpital, l'articulation services d'urgence-permanence de soins ambulatoires posent une vraie question.

Compte tenu du débat qui vient de se dérouler, je ne me fais aucune illusion sur le sort qui sera réservé à mon amendement ! Je propose tout simplement que les projets territoriaux de santé comportent systématiquement un volet portant sur la contribution des territoires aux formations des futurs praticiens.

personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Le projet territorial de santé est un outil de mise en cohérence de l'ensemble des projets des acteurs- que ce soient les projets des établissements de santé et médico-sociaux, des CPTS

Le conseil territorial de santé est composé de représentants des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie, ce qui permet de veiller à à articuler les projets territoriaux de santé avec les schémas départementaux des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.

Il nous semble en effet cohérent d'avoir une politique territoriale de santé qui tienne compte des diverses questions relatives à la politique départementale en matière d'accompagnement à domicile, de soutien aux aidants, de mobilité et d'accès au droit. L'amendement

pas utile de préciser que le conseil territorial de santé donnera un avis sur le PTS et en assurera l'évaluation. Il est normal qu'il s'assure de sa bonne articulation avec les autres orientations fixées, comme en matière de handicap au travers des schémas départementaux. La commission demande donc le retrait de ces amendements

en veillant à ce qu'il n'y ait pas de zones blanches, de territoires ou de sujets non couverts. En soi, l'objectif est louable, mais il comporte, à nos yeux, une faille : en effet, les projets territoriaux de santé sont laissés à l'initiative des acteurs de terrain, comme cela a été souligné à de nombreuses reprises.

de situations, nous considérons que l'État, en l'occurrence l'ARS, doit être le garant de l'existence et de la mise en place de ces projets territoriaux de santé. C'est pourquoi nous proposons, en cas de carence, d'offrir la possibilité au directeur général de l'ARS de saisir le conseil territorial de santé afin d'élaborer un projet sur le territoire concerné.

donc une demande de retrait ; sinon, avis défavorable. Mme Laurence Cohen. Il est indispensable que le fruit des évaluations de chaque conseil territorial de santé soit présenté au niveau régional, de même qu'il nous paraît indispensable que la mise en oeuvre du projet régional de santé puisse être évaluée annuellement et

? La définition des missions de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, la CRSA, lui permet déjà de se saisir de toute question portant sur l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation de la politique de santé dans la région et dans les

En outre, en particulier en milieu rural, les biologistes pourraient être mis à contribution pour soutenir et structurer les CPTS, dont ils pourraient même constituer l'ossature. Ils sont en effet habitués à fédérer des activités locales de taille moyenne.

une CPTS « est composée de professionnels de santé regroupés, le cas échéant, sous la forme d'une ou de plusieurs équipes de soins primaires, d'acteurs assurant des soins de premier ou de deuxième recours

président du groupe du RDSE, a demandé le retrait de la proposition de loi relative à l'accès effectif et direct des petites et moyennes entreprises à la commande publique inscrite à l'ordre du jour de l'espace réservé à son groupe du jeudi 13 juin 2019.